La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point le procès verbal est adopté sous les réserves d'usage. Mes chers collègues. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunis le 22 mars sont consultables sur le site du Sénat. N'ont pas reçu d'observation et je considère ces conclusions comme adopté. Madame. La Première ministre. Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance et retransmise en Direct sur Public Sénat et notre site internet. Au nom du bureau du Sénat. Chacun sera attentif à observer des valeurs essentielles qui sont le respect. Des uns et des autres et respect du temps de parole. Je commence par donner la parole au président Claude Malhuret. Pour le groupe les indépendants République et Territoires. Merci monsieur le président. Les scènes de guerre civile qui se sont déroulées samedi à Sainte-, Soline ont scandalisé les Français. Des Cars de gendarmes en feu. Des hors de de Black blocs venus de toute l'Europe bottés casqués cagoulés armés de cocktails Molotov, de boules de pétanque, de couteaux de machettes et de mortiers. Cette ultra gauche européenne a fait de la France, son terrain de jeu favori car elle sait qu'elle y trouvera un relais politique. Le relais de ce qui explique qu'il faut transformer les révoltes en révolution par un score par un slogan radical tout conflictualités Le relais de ceux qui défilaient samedi avec leurs écharpes tricolores dans une manifestation interdite illégal et ultraviolente pistant les forces de l'ordre par des textos sous des hashtags tout cramé. Et c'est la guerre. Alors que depuis plusieurs semaines, les organisations syndicales défilent dans le calme et la responsabilité. Les émeutiers organise désormais partout des cortèges parallèle brûle les ordures et les kiosques les portes des mairies et les préfectures cassent les vitrines des commerçants saccagent les permanences des parlementaires, menace de mort, les jeunes enfants des députés frappe des mères dont les projets ne leur plaisent pas et en définitive finissent même par terroriser les manifestants pacifiques l'ultragauche pyromane se moque des retraites et les mégabassines. Son objectif c'est l'insurrection sa cible la République qu'elle est bien décidé à abattre pour faire de la France un nouveau Venezuela. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier à l'Assemblée. De premières sanctions contre certains des traînes savates incendiaire. Je voudrais que vous nous assuriez madame, la Première ministre, que votre gouvernement prendra toutes les mesures politiques réglementaires judiciaires pour protéger ceux qui nous protègent, policiers, gendarmes, pompiers, élus et plus généralement toutes ces personnes menacées par ces factieux. Les forces de l'ordre ont eu au cours des dernières semaines plus de 400 blessés dont 47 ce week-end à Sainte-, Soline. C'est à ce prix qu'elle nous protège et je voudrais qu'ici c'est la moindre des choses. Nous leur rendions hommage par nos applaudissements.

Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le président, Claude Malhuret. Comme vous et comme bon nombre de nos compatriotes. J'ai été profondément choqué par le déchaînement de violence ce samedi à Sainte-, Soline contre les gendarmes. Contre l'ordre républicain. J'ai été choqué de voir des élus se rendre en écharpe tricolore à une manifestation interdite. J'ai été choqué ces dernières semaines d'entendre des élus multiplié les propos incendiaires et parfois même justifié les violences. Renvoyer dos à dos casseurs et forces de l'ordre. C'est indigne de la part d'élus de la République. Alors aujourd'hui avec vous avec les Français, je veux à mon tour, rendre hommage aux forces de l'ordre à leur courage et à leur engagement. Je veux dire ma solidarité aux gendarmes et aux policiers qui qui ont été blessés à Sainte-, Soline ou dans les débordements qui ont malheureusement parfois entouré les mobilisations ces derniers jours. Mesdames, et messieurs les sénateurs, hein. Les policiers et les gendarmes connaissent leur devoir d'exemplarité et de respect de la déontologie le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, l'a encore rappelé hier. Des casseurs et des militants radicalisés venus chercher l'affrontement et défier nos institutions sont à l'origine des scènes que nous avons vu ces, ces derniers jours, notamment à Sainte-, Soline c'est leur comportement qui mettent en danger chacun, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, secours et même les manifestants. Alors, de notre côté, nous faisons tout pour éviter que des débordements surviennent et comme vous tous ici, j'ai une pensée pour les deux manifestants toujours hospitalisé dans un état très grave. Depuis samedi. Depuis des semaines. Le ministre de l'Intérieur, les préfets, les forces de l'ordre au contact des organisations syndicales travaillent ensemble et ont permis la tenue de la grande majorité des mobilisations sans heurts. Nous continuerons à nous adapter et à réagir pour que la violence ne supplante jamais l'expression des revendications. C'est le sens du dispositif qui encadrer la journée d'hier, il a permis d'éviter de nombreux débordements affrontements dégradation. C'est le sens de la procédure de dissolution annoncée hier par le ministre de l'intérieur du groupuscule soulèvements de la Terre, mesdames et messieurs les sénateurs. La violence n'a pas sa place dans les cortèges et nous sommes déterminés à continuer à protéger tous ceux qui veulent exprimer pacifiquement leurs idées à protéger les Françaises et les Français. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Daniel crémier pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président. Madame, la Première ministre Madame et messieurs les les ministres chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre. Ce qui vient de se passer de. Autour de la retenue d'eau de Sainte-, Soline dans mon département des Deux-Sèvres a bouleversé la France entière. Sainte-, Soline c'est 357 habitants qui viennent de vivre en moins de six mois un second état de siège. Je tiens à dire à ses 357 habitants. Toute ma compassion ma compassion et mon total soutien ainsi qu'aux agriculteurs et aux gendarmes. À quoi avons-nous assisté samedi dernier devant nos écrans de télévision. Certainement pas une manifestation ordinaire d'ailleurs interdite par la préfète du département. Vous avez vu des centaines de casseurs armés organisée rompu à l'exercice est déterminé à faire reculer l'État en cassant du gendarme. Avec un bilan redoutable des dizaines de blessés chez les gendarmes et les manifestants, mais aussi avec le soutien d'élus de la République qui se trouvait sur le terrain, c'est intolérable. Monsieur le Ministre, comment en sommes-nous arrivés là. Comment expliquer qu'en France, en 2023 on puisse être confronté à une telle violence à intervalles réguliers. Le sujet n'est plus celui de l'eau et pas davantage celui de l'agriculture, le sujet c'est l'autorité de l'État. Alors Monsieur le Ministre quand l'extrême violence semble habituel dans ces rassemblements. Qu'entendez-vous faire pour restaurer l'autorité de l'État et mettre un terme à l'activisme des casseurs qui servit qui sévissent dans les manifestations. Pour vous répondre. La parole est au ministre de l'Intérieur, les Outre-mer monsieur Gérald Darmanin. dire tout mon soutien aux habitants de votre département a singulièrement à ceux de Sainte-, Soline mais également aux agriculteurs. Parce que café l'état pendant deux week-ends de suite qu'ont fait les gendarmes puisque si nous comptons les deux week-ends affrontements c'est plus de 100 gendarmes qui ont été blessés, parfois très gravement que de protéger l'outil de travail des agriculteurs que de protéger ses agriculteurs des Deux-Sèvres, mais partout en France qui sont parfois l'objet de menaces d'intimidation d'insultes de la part de gens qui utilisent en effet la violence verbale et physique pour arriver à leurs fins politiques. Monsieur le sénateur, le ministre de l'Intérieur applique le droit à l'et la loi de la République, il n'a pas la possibilité d'interpeller les gens avant que des faits se soit commis même lorsqu'ils sont connus par les services de renseignement. Je voudrais rappeler d'ailleurs ici que la proposition de loi de monsieur Retailleau qui a été reprise par mon prédécesseur a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel qui empêche le ministre de l'Intérieur qui ne fait qu'appliquer le droit dans un état droit et de constater les infractions avant de éventuellement pouvoir interpeller ces personnes constatons d'ailleurs que lorsque le ministre de l'Intérieur fait procéder à ces interpellations, il est lui-même critiqué mais c'est un autre sujet. Il vaut mieux critiquer mise intérieur que les que vomir sur les policiers, gendarmes, comme l'a fait une partie de la de gauche et d'extrême gauche ces derniers jours le 2ème. Sujet, monsieur le sénateur, c'est qu'il faut faire voler des drone trois avoir des images, qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-, Soline. Les casseurs ont pu faire voler des drone pour regarder le dispositif des gendarmes et les policiers, les gendarmes vous avez refusé mesdames et messieurs les drone pour les policiers, gendarmes, sont les seuls. À ne pas pouvoir faire voler des drone. Alors oui, il faut en tirer toutes les conclusions. Je veux quand même souligner le travail de nos gendarmes courageux, il n'y a pas eu de Zad à Sainte-, Soline pendant deux week-affrontements et c'est aussi ça l'autorité de l'État. J'ai remercié les gendarmes. Monsieur le Ministre. Mais posons-nous la question. J'ai pris note des explications que vous m'avez donné mais je crois que nous sommes dans une ère nouvelle qui a commencé avec la reculade de l'État à Notre-Dame des Landes.

La parole est à notre collègue Jean-Pierre Moga, pour le groupe de l'Union centriste. Merci, merci, Monsieur le président, Monsieur le Ministre samedi dernier plus de 80 maires et de nombreux habitants manifesté devant le pôle de santé du Villeneuvois contre le risque de fermeture de la maternité. En effet, en Lot-et-Garonne, comme dans de nombreuses autres départements ruraux d'outre-mer ou en Corse. L'entrée en application de la loi Rist. Le 3 avril aura pour effet de bord inéluctable une réduction, voire la fermeture de services d'urgences et de maternité dans les hôpitaux. Comme vous le savez, le maintien de ces services publics essentiels constituent un enjeu majeur pour la santé et pour les territoires concernés. Les femmes enceintes sont souvent contraintes de parcourir de longues distances pour accéder à l'hôpital le plus proche. Ne pas avoir la certitude de pouvoir accoucher à proximité de son domicile est extrêmement anxiogène. Nous sommes en droit d'attendre de votre part une réponse qui dépasse les logiques comptables à l'origine de la dégradation des services. Je partage l'objectif fondamental de plafonner la rémunération de l'intérim médical qui s'apparente dans certains cas. Sont à un chantage exercé sur le service public de la santé, au mépris des principes humanistes de la médecine. En revanche. L'application de cette loi peut avoir des effets catastrophiques sur nos petits hôpitaux. Monsieur le Ministre. Pensez-vous que les habitants des zones rurales sont des citoyens de seconde zone. Quel signal comptez-vous leur envoyer dans les prochains jours. Monsieur le ministre, quelles mesures urgentes envisagez-vous de prendre afin de préserver en priorité nos maternités rurales et nos services hospitaliers. avez-vous l'intention d'abaisser en zone rurale. Le seuil de 1000 naissances par an afin d'y maintenir la maternité je vous remercie.

il y a bien entendu pas de citoyens de seconde zone et mon travail sous l'autorité de la Première ministre, c'est de rétablir l'accès à la santé équitable pour tous sur l'ensemble de nos territoires. Vous évoquez de problèmes le 1er concernant l'intérim médical mais nous parlons bien ici des dérives de cet intérim médical et non de l'intérim qui est qui est normal et y'qui fonctionne et qui permet de maintenir justement ces ces petites structures ces dérives d'intérim médical. Elles sont à court terme, soyez-en certain. La mort de notre service public hospitalier quel médecin acceptera encore de travailler pour 4000 euros par mois. Lorsqu'un intérimaire venant 24h aura la même somme. Par rapport à, à ces dérives de l'intérim médical, il faut agir sur les 2 tableaux lutter contre les dérives et aussi préserver cette colonne vertébrale de notre système public hospitalier que sont les médecins hospitaliers. C'est pourquoi nous agissons des deux côtés. Tout d'abord la limitation de l'intérim, vous l'avez dit, ensuite favoriser l'exercice des médecins hospitaliers en prolongeant les mesures de cet été. Ces mesures qui permettent d'augmenter la rémunération pour les gardes de nuit à le week-end de reconnaître la pénibilité. Également en développant ce qu'on appelle la prime de solidarité territoriale qui permet. À un médecin hospitalier d'aller aider dans un autre hôpital elle devient très intéressant aussi financièrement. Enfin nous avons relever ce plafond de l'intérim. Il avait été défini en 2016 avec les évolutions depuis est maintenant à 1390 euros brut par mois. Concernant les petites maternités, vous évoquez par la notion de 1000 naissances, le rapport du professeur Yves Ville, rapport qui l'a fait à la demande et à l'Académie de médecine. C'est un rapport fait par des scientifiques, c'est un rapport scientifique qui n'engagent en aucun cas bien entendu le gouvernement ni mon ministère, je vous rejoins dans la volonté de maintenir ces unités de proximité mais nous devons aussi réussir à combiner sécurité qualité et proximité. C'est ce à quoi je m'y emploie. Je vous remercie. La parole est à d'autres collègues Fabien Gay pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste avait la parole. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre depuis une semaine le débat public se concentre sur les violences dans les manifestations. Retraites, elles doivent être condamnés sans ambiguïté mais elles ne peuvent détourner l'attention des vraies questions. La vraie question c'est qu'après 3 mois de mobilisation. Une majorité de Français refusent toujours de travailler 2 ans de plus pour satisfaire les marchés financiers. La vraie question c'est qu'après votre passage en force au Parlement en détournant des moyens constitutionnels ventre légitimité démocratique est considérablement affaibli. La vraie question c'est la répression syndicale et les réquisitions. La répression du mouvement social avec des NAS pourtant interdite, des arrestations arbitraires des armes offensives qui blesse et doivent être proscrites et la violence policière de la BRAV M révélés par des enregistrements parus dans la presse et qui doit être dissoute. La vraie question c'est que vous avez perdu toute autorité politique que vous êtes seul et que vous ne renouerait pas avec le pays en restant confinés. La vraie question c'est qu'hier vous railler une foule mais c'est un fait. Un peuple qui se tient devant vous droit digne, fier, calme et qui avec le mouvement social uni et rassemblé veut être respecté entendu madame, la Première ministre en politique il faut avoir des convictions et les a affirmé parfois contre vents et marées. Mais lorsque vous piétiner la démocratie sociale, lorsque vous humilier le Parlement lorsque vous risquez des drames par le choix de l'autoritarisme. C'est le signe qu'il ne faut pas s'entêter l'audace en politique c'est parfois reconnaître qu'on a eu tort et renoncer. Notre pays a besoin de sortir de la crise sociale, politique et démocratique dans laquelle vous l'avez plongé. C'est le seul apaisement possible et il doit venir de vous. Nous vous proposons 2 issue politique. Le retrait de la réforme ou le référendum d'initiative partagée. Madame, la Première ministre allez-vous enfin écouté et respecté la majorité du peuple français. majorité du peuple français. Monsieur le ministre du Travail, monsieur Dussopt, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur gay vous interroger madame, la Première ministre et le gouvernement sur. La mise en oeuvre que vous contestez de la réforme des retraites. Je voudrais d'abord revenir, monsieur le sénateur, mais ce sont des arguments. J'ai déjà partagé avec vous sur le fait que ce projet de loi et d'abord la concrétisation d'un engagement pris par le président de la République et par les candidats de la majorité présidentielle aux élections législatives, que nous avons conduit avec la Première ministre. Quatre mois de concertation et qu'à l'issue des 4 mois de concertation. Le texte a été considérablement enrichi sur des questions de prévention de l'usure professionnelle sur des questions des prix des questions relatives aux carrières longues ou encore au minimum de pension. Nous avons aussi mis à profit le débat parlementaire. Ce sont 175 heures de débat parlementaire. C'est plus que l'addition des 2 réformes précédentes 175 heures qui ont permis là aussi d'enrichir le texte et de l'enrichir considérablement. Monsieur le sénateur, vous dites. 2 choses à l'occasion de votre question, la première c'est que vous vous et je partage vous condamner les violences qui sont commises en marge des manifestations et c'est une manière je crois toujours, vous l'avez dit, c'est une manière je crois de, de partager l'hommage régulièrement rendus par le gouvernement et singulièrement par le ministre de l'Intérieur à l'action des forces de police pour protéger les cortèges et garantir le maintien de l'ordre et ensuite monsieur le sénateur, vous dites, nous vous proposons de 2 issus le référendum ou le retrait du texte. Permettez-nous d'en emprunter une troisième la troisième c'est celle du dialogue social et de la reprise du dialogue. C'est la raison pour laquelle la Première ministre a proposé à l'intersyndicale de les recevoir dès le début de la semaine prochaine pour travailler sur les sujets d'usure professionnelle de déroulement de carrière de bien notre travail, c'est la raison pour laquelle aussi, monsieur le sénateur, nous souhaitons que l'ensemble des initiatives prises par les partenaires sociaux, je pense notamment à l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur puisse aussi faire l'objet de de concertation de travail commun pour qu'il puisse être on faisait pas la loi, le dialogue, toujours le dialogue, et des portes toujours ouvertes pour faire en sorte que nous puissions avancer. La parole est maintenant à notre collègue Marie-, Laure Phinéra, or pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre samedi dernier la Guyane s'est réveillé sous le choc. Arnaud blanc maréchal des logis-chef de l'antenne locale du GIGN a été tué lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Nos pensées d'ailleurs vont à sa famille, ses proches ainsi qu'à ses frères d'armes. Ce drame intervient quelques jours après que des hommes armés de mitrailleuses Kalachnikov ont braqué un autre site d'orpaillage et ont pris en otage le personnel et un pilote d'hélicoptère. Ces incidents sur les conséquences d'une forte augmentation de l'orpaillage illégal mais aussi de la présence de factions en provenance du Brésil. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. En effet, depuis son investiture, le président Lula, a déclaré la guerre à l'orpaillage clandestin au Brésil ainsi près de 20.000 garimpeiros ont été chassés de la réserve Yanomami. On estime à 5000 le nombre d'empailleur illégaux qui pourrait ainsi rejoindre la Guyane est porté à 11.000 le contingent de chercheurs d'or illégaux sur notre territoire pour ne rien arranger, sur les marchés internationaux le cours de l'or ne cesse de s'envoler. Ces dernières semaines. Dans les sous-sols de la Guyane plus attractif que jamais. Vous connaissez monsieur le Ministre des enjeux environnementaux et sécuritaires auxquels est confrontée la Guyane en 2017, le président de la République lui-même avait conditionné nos aides et nos relations diplomatiques avec le Brésil et le Suriname à une coopération policière et judiciaire contre l'orpaillage illégal. 6 ans plus tard et malgré les opérations Harpie l'orpaillage illégal demeure un fléau hors de contrôle. C'est pourquoi monsieur le ministre, je souhaiterais connaître précisément les mesures que vous entendez prendre pour intensifier l'action de l'État en matière de lutte contre l'orpaillage illégal préserver l'intégrité du territoire guyanais protéger les populations guyanaises et préserver l'environnement. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, ce sénateur madame la sénatrice, merci et je veux avoir comme vous au nom de la Première ministre et du gouvernement. Une pensée pour la famille. Et et pour. Le sacrifice du maréchal et le. Logis-chef blanc militaires du GIGN très rompu à l'exercice et qui a trouvé effectivement la mort sans doute assassiné, l'enquête le dira par ce que vous dénoncez. Permettez moi aussi d'avoir une pensée pour les, les sapeurs-pompiers de Paris qui. Connaissent au moment où je parle un accident extrêmement grave de la route en Guyane là aussi avec plusieurs pronostic vital engagé. Je sais que je parle au nom de la représentation nationale en associant évidemment. À. Je veux dire madame la sénatrice, que la lutte de la France. Contre l'orpaillage illégal est une lutte pour la souveraineté. Bien sûr une lutte contre les trafics de tous genres et une lutte contre l'insécurité qui touche nos compatriotes guyanais. Vous l'avez dit vous-même ces bandes armées qui pillent le sol de la Guyane, qui pollue parce que c'est la protection de l'environnement qui est évidemment en jeu mais qui ensuite revendent et ensuite vont dans les villes de Guyane hé bien sûr à Cayenne, mais pas simplement faut aussi naître les augmentations d'homicides et de tentatives d'homicide que votre collectivité connaît depuis trop longtemps. Alors le gouvernement a augmenté les moyens, 250 policiers et gendarmes depuis 6 ans. L'opération Harpie civilo-militaire gendarmerie nationale mais également de l'armée, je parle aussi au nom bien sûr de bien sûr de Sébastien Lecornu a été renouvelé ce le président Hollande parce qu'elle avait été imaginé en 2008 et renouvelé ce président Macron en 2018 et je sais qu'autour de la Première ministre nous réfléchissons à renforcer des moyens notamment militaires. Dans le cas de la loi de programmation militaire qui vous sera bientôt proposée pour prendre en compte le nouveau deal brésilien que vous évoquez la protection de la plus grande frontière qu'à la France hein. Qu'un pays étranger, c'est-à-dire le Brésil évidemment tenir la protection de la forêt amazonienne avec toutes les difficultés que nous connaissons le sacrifice. Du militaires du GIGN ne n'est pas vain. Il est évidemment comme tous ses autres camarades. Un soldat de la protection de nos frontières de nos compatriotes guyanais, ce n'est pas simplement pour protéger une forêt c'est déjà beaucoup les militaires du GIGN sont dans la forêt amazonienne en Guyane c'est pour protéger évidemment les Guyanais des règlements de compte extrêmement nombreux que nous connaissons depuis de trop nombreux moi. Merci. La parole est maintenant au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste écologiste. Monsieur Monsieur le président, madame, la Première ministre. J'ai regardé attentivement les dernières déclarations qui pouvait définir votre ligne politique depuis l'échec de la réforme des retraites entérinée par votre absence de majorité sur ce texte. Je retiens le ni dissolution ni remaniement ni référendum du président de la république et votre proposition de dialoguer la semaine prochaine avec les syndicats, mais sur les seuls sujets sur lesquels vous êtes d'accord, selon les mots mêmes de votre ministre Franck Riester. On vous mettant au service d'un président de la République du triple ni pour ne pas dire du déni. Vous êtes devenu la première Ministre de l'impasse. Malgré toutes vos tentatives de diversion malgré votre stratégie assumée du pourrissement. L'opposition à votre réforme des retraites n'a jamais été aussi massive. Parmi les Français. Le mouvement social et le plus important depuis des années 90, les syndicats montrent depuis le début de cette mobilisation leur grande responsabilité en les traitant comme vous le faites, madame, la Première ministre. Vous jouez avec notre pacte républicain. Je ne veux pas que vous noyer le poisson, le poisson en assénant au Sénat vos habituels éléments de langage sur une réforme dite indispensable pour sauver notre système de retraite, plus personne ne vous croit. Et si vous évoquez l'actuel climat de violence inacceptable qui a émaillé certaines manifestations avec les syndicats. Nous les avons dénoncé comme nous l'avons toujours fait et nous aussi, mes chers collègues, nous soutenons l'ordre républicain et ceux qui le défendent. Policiers et Jean. Armes. droit, nous avons le droit. D'interroger la doctrine du maintien de l'ordre du gouvernement l'espèce, ce que je veux madame, la Première ministre, c'est que vous répondiez à la proposition de l'intersyndicale que vous acceptiez la médiation que vous suspendez l'application de cette réforme injuste et inutile que vous preniez en compte la réalité, il n'est plus tant de jouer avec les matamores le jouer les matamores comme le fait Emmanuel Macron. Il est temps de répondre avec sérieux aux demandes des syndicats. Je vous offre une tribune profitez en. en. Répondent. La parole est à madame la Première ministre. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Patrick Kanner. Comme chacun ici. Qu'il se soit opposé à la réforme des retraites ou qu'il ait voté. Je vais au contact des Français. J'entends leurs craintes, leurs espoirs et parfois leur colère. Comme chacun ici j'entends les revendications de celles et ceux qui prennent part au mouvement social. Des revendications qui dépassent la réforme des retraites. Comme chacun ici je suis attentive aux témoignages des élus locaux qui sont en première ligne face aux difficultés de nos concitoyens. Comme chacun ici je connais les attentes des Français pour leur pouvoir d'achat pour leur santé, pour l'éducation de leurs enfants. Alors Monsieur le Président can ma conviction aujourd'hui c'est qu'il ne faut pas chercher à renforcer les craintes qu'il ne faut pas chercher à attiser les colères. Aujourd'hui il faut apaiser le pays en rassemblant les bonnes volontés. Toutes celles et ceux au delà des clivages qui sont prêts à trouver des solutions. Aujourd'hui, il ne faut pas renoncer à agir. Au contraire, il faut accélérer apporter des réponses concrètes qui améliore le quotidien des Françaises et des Français. C'est aujourd'hui autour de ces 2 axes, ce que je souhaite bâtir dans les prochaines semaines un programme de gouvernement et un agenda législatif comme le président de la République m'en a confié la tâche depuis lundi. J'ai donc entamé une série de consultations. J'ai vu hier le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Je l'ai poursuit avec les forces politiques, les parlementaires, les élus locaux et les partenaires sociaux, que j'ai envie inviter à une rencontre en début de semaine prochaine. Ma seule ambition, c'est de trouver des solutions au service des Français et de bâtir des majorités de projet pour les mettre en oeuvre toutes celles et ceux qui veulent agir pour les Français sont les bienvenues. C'est de cette manière par la concertation, par le dialogue et par le compromis que nous répondons répondront aux inquiétudes de nos compatriotes. Je vous remercie. Monsieur le président. Programme de gouvernement nous répond Madame Élisabeth Borne. Mais madame Borne. Ça fait 70 mois. 70 moi que vous êtes au pouvoir avec vos amis politiques vous n'avez plus de boussole et surtout je le pense très sincèrement, vous ne comprenez plus l'esprit des Français et c'est ça qui est terrible aujourd'hui dans notre pays. La parole est à madame la présidente Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, vous avez la parole. Merci, merci monsieur le président, madame, la Première ministre, Monsieur le Ministre de la Santé. Mes chers collègues. Notre jeunesse, c'est en grande souffrance psychologique. De plus en plus de jeunes font face à un état dépressif et certains vont jusqu'à intenter à leurs jours, et nous les pleurons un à. Pression sociale pression des réseaux sociaux harcèlement éco-anxiété crise sanitaire, les crises de ce mal-être sont multifactorielles les cons les séquences terrible. Le Haut Conseil de la famille de l'enfance et de l'âge, vient de publier un rapport intitulé quand les enfants vont mal comment les aider. Les chiffres concernant la consommation médicamenteuse sont glaçants. Chez les 6 17 ans, un jeune sur deux consomment des psychotropes. En 8 ans, cette consommation a explosé. Plus 49% d'antipsychotiques, plus 55% d'hypnotiques et sédatifs, plus 63% d'antidépresseurs. Ce phénomène de sur-médication ne concerne pas des cas isolés mais bien des dizaines de milliers d'enfants et place la France parmi les pays les plus prescripteurs des médicaments qui plus est pour adultes car aucune médication de ce type n'est autorisé sur le marché aujourd'hui pour nos enfants. La France privilégie donc le traitement des symptômes puisqu'elle est sous-dotée des capacités à agir sur les racines du mal. Car là est le coeur du problème, la psychiatrie, le parent pauvre de la médecine. Nous comptons seulement 600 pédopsychiatre pour près de 10 millions d'enfants. La Cour des comptes préconise d'ailleurs de dresser l'état des lieux de cette spécialité. 800 médecins scolaires soit un médecin pour 15.000 élèves. Imaginez-vous l'état de désemparement des parents qui se battent corps et âme pour permettre à leurs enfants d'avoir une Systems s'psychologique quand on leur annonce que pour obtenir une place dans un centre médico-pédagogique, il faut attendre 2 ans. La France elle aussi attend depuis des années son plan psychiatrie financer madame, la Première ministre monsieur Fiole Ministre de la Santé. Il est grand temps d'établir ce plan budgétaire et doser érigé la psychiatrie en grande cause nationale. Je vous remercie. Pour vous répondre. La parole est au ministre de la Santé et de la prévention. La santé mentale est une priorité, bien entendu et la santé mentale des jeunes encore plus pour ce gouvernement et que je partage avec mes collègues Pap Ndiaye Sarah El Haïry et Charlotte Caubel, bien entendu. Nous n'ignorons rien des difficultés de la pédopsychiatrie difficultés qui ne sont pas nouvelles, vous avez rappelé le chiffre des des pédopsychiatres qui est bien insuffisant. Mais je vous le rappelle qu'il faut 10 ans pour former un médecin, ça va être long. On va pas régler le problème tout de suite pour autant nous agissons quand même nous agissons depuis la feuille de route qui a été mis en place en 2018, renforcée en 2021 par les Assises de la santé mentale, qu'est-ce qui a été fait déjà le. Le programme des 1000 premiers jours qui permet un accompagnement ensuite la mise en place des maisons des adolescents il y a maintenant une maison des adolescents au minimum dans chaque département il y a également des structures qui se déploient pour aller vers les jeunes dans nos zones rurales qui sont le plus loin des des grandes villes, c'est en particulier le cas à Poitiers avec un bus qui se déplace avec une équipe de la Maison des adolescents. Et puis il y a également le déploiement de mon parcours psy. On dit beaucoup de choses sur mon parcours psy mais avec plus de 300.000 consultations depuis que cela a été créée, dont 20% pour des jeunes mineurs. C'est un véritable succès sur lequel il faut que nous construisions aussi l'avenir. J'attends dans les prochaines semaines les conclusions des assises de la santé de l'enfant et de la pédiatrie que j'ai lancé pendant la crise de cet hiver dans ces assises il y a un des 6 chapitres qui est entièrement consacré à la pédopsychiatrie, nous aurons à construire ensemble et à échanger sur la feuille de route pour la pédopsychiatrie des prochaines années. Je vous remercie.

Et je l'assume. De manifestants dans le coma entre la vie et la mort de ton espère une sortie sans séquelles graves, 47 blessés parmi les forces de l'ordre à qui nous souhaitons évidemment un prompt rétablissement. 200 blessés dont certains mutilés. Parmi les manifestants à qui nous souhaitons aussi un prompt rétablissement des violences inqualifiables se sont déchaînés et nous les dénonçons toutes sans ambiguïté mais c'est votre bilan du week-. Monsieur le Ministre, vous avez décidé à Sainte-, Soline d'exposer 3000 forces de l'ordre à la violence dans un Champ pour défendre quoi qu'il en coûte un trou, un trou vide vous avez décidé d'interdire une manifestation totalement légitime parce que vous êtes incapables de faire respecter la loi en matière de partage de l'eau. Oui, de nombreuses bassine déclarées illégales sont toujours en construction et vous êtes incapable d'assumer votre responsabilité oui la bassine de Sainte-, Soline met en danger la ressource en eau de tout le territoire depuis 3 jours. Vos mensonges ont éclaté au grand jour des armes de guerre ont bien été employé samedi des brigades motorisées était bien équipé de LBD. Des secours ont été entravés. Et empêcher d'intervenir sur hors de la gendarmerie des gaz lacrymogènes ont été envoyées sur des sur vous mentez comme vous avez monté ici lors du fiasco du Stade de France. Dans quel pays. Après avoir mis de manifestants dans le coma. Toute la chaîne de commandement ne s'interroge pas sur la méthode de maintien de l'ordre dans quel pays après un tel fiasco. Un ministre peut continuer de mentir à répétition et peut dissoudre un collectif d'opposants politiques. Merci monsieur le président vous avez su les sénateurs parce que 16h. Je n'ai pas. Tout compris de votre question. Vous, oui il y avait un peu de bruit mais je crois que vous faisiez une différence entre la gauche et le gauchisme finalement dans votre intervention et je regrette que des parlementaires au revendique d'aller dans une manifestation illégale. Ne respectant ainsi pas eux-mêmes la loi de la République. Je regrette que des parlementaires puissent être à côté de ceux qui jettent des cocktails Molotov sur des gendarmes. Je regrette. Que des parlementaires puissent ne pas constater comme j'ai pu le constater de voir des gendarmes dont les pieds eux- mêmes ont été attaqués par l'acide. Je regrette monsieur le sénateur que vous n'ayez pas entendu les deux conférences fait de conférence de presse faites par Madame la préfète avant la manifestation, qui était interdite depuis le 17 mars, ni même celle du procureur de la République manifestement vous êtes assis sur tout ça. Sur les violences contre nos gendarmes sur l'interdiction de manifestation sur les conférences de la préfète de la République sur la conférence du procureur de la République je regrette par ailleurs que vous relayez ici de nouveaux défectueuse. Non monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Oui monsieur mais écoutez le SAMU regarder le SAMU, le SAMU des Deux-Sèvres qui le dit lui-même je sais que ça vous ferait plaisir de penser que gendarme souhaite la mort des gens. Mais ce n'est pas le cas. C'est le médecin du GIGN. Monsieur le sénateur qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par manifestement vos camarades d'un jour. Mais vous pouvez hocher la tête c'est extrêmement scandaleux ce qui se passe les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour parce qu'alors qu'il allait secourir un manifestant. Il se faisait harceler par des pluies de pavés et de cocktails Molotov. Voilà la vérité. Monsieur le sénateur. Et moi aussi je vais avoir une pensée bien sûr pour toute personne qui a été blessées manifestement pour ceux qui luttent pour la vie et l'enquête judiciaire dira ce qu'elle dira la vérité et je suis évidemment prêt avec tous les administrations pour lui répondre, j'ai dit au président de la commission des lois que j'étais à sa disposition comme à l'Assemblée nationale pour répondre à vos questions. Mais il y a un truc, il y a une chose, vous. Il y a une chose Monsieur président pardon je ne ferai pas s'est crashé comme vous le faites sur la tête des forces de l'ordre.

Vous ne pourrez pas organiser une manifestation à huis clos. Vous ne pourrez pas épargné à huis clos. Mais vous êtes le ministre d'un pays où le président ne peut plus sortir de son palais. Vous êtes le ministre d'un gouvernement, il faut compter tout présentée comme celle d'un contrôle du Parlement. Vous êtes le ministère public ont pu bloquer fracturé par votre les tarifs. Vous comptez terminé. De la parole est à madame Le Laurence Garnier pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Olivier Véran, ministre en charge du renouveau démocratique. Monsieur le Ministre, en 2021 les violences contre les maires et les élus ont augmenté de 47%. En 2022, elles ont à nouveau augmenté de 32%, donc en 2 ans. Ces violences ont presque doublé. Alors il s'agit d'insultes, d'agressions mais aussi désormais d'actes criminels. La semaine dernière la voiture et la maison du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique ont été touchées par un incendie volontaire. Monsieur le Ministre ces violences. Seuls leurs auteurs en sont responsables. Mais les élus locaux paye aujourd'hui un climat de défiance que vous avez contribué à aggraver je rappelle qu'en 2018 l'actuel ministre de l'Intérieur a publié la liste des maires augmentant la taxe d'habitation. S'en est suivi la campagne de dénigrement. BalanceTonMaire orchestré par les militants de votre mouvement politique. Monsieur le Ministre. Vous semblez avoir aujourd'hui pris la mesure de la situation les mesures et des derniers textes de loi adoptés vont dans le bon sens mais le remède court après le mal de nombreuses plaintes reste classée sans suite. Les agressions se poursuivent. Souvent dans la plus grande impunité. Monsieur le Ministre, avant de vous lancer dans le renouveau démocratique dont vous avez la charge, comment allez vous protéger ceux qui font vivre notre République au quotidien dans les 35.000 communes de France. Pour vous répondre. La parole est au ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Laurence Garnier. Je vous remercie de m'interpeller comme Ministre délégué chargé du renouveau démocratique au sujet des violences dont sont victimes de plus souvent et de plus en plus en plus souvent les, les élus de la République. Il faut dire d'abord, je partage votre émotion et votre colère face à des actes de violence qui s'accentue et qui devient de plus en plus nombreux. On va avoir une divergence sur le diagnostic, madame la sénatrice, parce que quand on regarde l'histoire, histoire contemporaine française mais aussi l'histoire occidentale en général. On voit que les élus commencent à être pris pour cibles par les populations lorsqu'elles sont en colère, depuis une vingtaine d'années en réalité et il y a un phénomène qui, qui tend à s'accroître. Madame c'est la on peut y voir plusieurs continuum probablement une forme de continuum entre la violence anonyme et sans conséquence des réseaux sociaux et la violence qui peut s'exprimer dans la rue ou lors de conseils municipaux. On peut y voir un continuum entre la violence qui parfois s'exprime au sein même de la maison du peuple au sein même du Parlement je parle. Essentiellement de l'Assemblée nationale, on l'a vu au cours des dernières semaines et la violence qui peut s'exprimer dans la rue. Nous devons faire figure d'exemple, nous devons faire bloc pour montrer aux Français que si nous pouvons partager des divergences idéologiques profondes, si nous pouvons être en désaccord profond sur certaines lois certaines mesures en aucun cas nous ne perdons le respect de l'autre, en aucun cas nous ne perdons l'estime pour l'autre. Madame la sénatrice. Il se trouve que j'ai contacté quelques heures après l'incendie. Le maire Yannick mauresque est le maire de. Saint-Brévin-les-Pins parce que j'avais été profondément émue de constater alors il, il y aura une enquête pour pouvoir le démontrer mais que du simple fait qu'il ait accepté la mise en place d'un centre d'accueil pour réfugiés à la demande d'ailleurs de l'État et c'est son rôle, de l'accepter, il a été d'abord victime de menaces de mort d'injures puis finalement a vu son domicile dégradée avec la l'incendie c'est de voitures et dégradation d'une partie de sa maison par vous dites par qui. Madame la sénatrice.

ou de droite, l'ultra-droite et l'ultra-gauche sont les ennemis que nous combattons et que nous devons combattre et vous ne verrez jamais d'ambiguïté. Vous ne verrez jamais d'ambivalence et vous ne verrez jamais de oui mais lorsqu'il s'agit de condamner des violences retirer Lemay retirer le mais après le. Hé oui et ensuite vous aurez des leçons madame la sénatrice, madame la sénatrice, pour terminer, vous dire que nous devons faire ce travail pédagogique, il pourra l'expliquer aux populations. Pour protéger les mères. Ils font partie la la nation et s'attaquer un maire, c'est s'attaquer la vous conclut-elle vous plongera les siens. Madame Garnier vous avez quelques secondes. Oui, merci Monsieur le Ministre pour vos réponses ce, ce qu'on voit tous c'est que les Français votent de moins en moins et que les élus se font agresser de plus en plus, donc je crois effectivement que nous devons tous ensemble résoudre cette crise démocratique que nous traversons. Si. La parole est à madame Marie-. Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le président, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Tout le monde ici condamne les violences d'où qu'elles viennent et quelles qu'en soient les victimes. Manifestants et forces de l'ordre dont nous avons salué l'engagement nous le Stallion encore à l'instant. C'est pourquoi les faits commis par la brave la semaine dernière à Paris sont inacceptables. Valentin, 19 ans, je suis projeté au sol une moto me roule sur la jambe gauche hématome de 56 centimètres Sulayman 23 ans tu as tellement de chance d'être assis là je te jure je te péter les jambes au sens propre, je peux te dire qu'on en a cassé des coups des des gueules Salomé, 22 ans ta vie ne tient qu'à un fil. Je vois la peur dans ton regard j'aime ça. Paul Boyer, journaliste, 25 ans, sans un mot, un agent de la BRAV, le frappe au visage, avec une matraque traumatisme crânien, fracture de la main gauche. vous engagez-vous ici aujourd'hui a adressé à l'ensemble des forces de l'ordre. La lettre du 29 mai 1968 de Maurice Grimaud, préfet de police de Paris qui disait, nous n'avons pas le droit de passer sous silence les excès dans l'emploi de la force. Frapper un manifestant à terre c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière, vous devez faire une guerre impitoyable à tous ceux qui par leurs actes inconsidérés accréditerait l'image déplaisante, que l'on cherche à donner de nous. On vous répond la parole et ministre de l'intérieur des Outre-mer. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs, 7h, madame la sénatrice. Qui est comme dans toute profession comme dans toute activité des policiers, des gendarmes qui ne respectent pas les valeurs le droit, la déontologie, c'est une évidence. Et d'ailleurs j'en ai sanctionné. Plus que la moyenne. Lorsque vous étiez aux responsabilités le quinquennat d'avant. Vous avez connu des périodes où les manifestations ont été difficiles, je pense à la loi travail de matériel connerie ou des difficultés de match à de lourdes je pense à Sivens que vous citez peu finalement dernièrement dans les interventions du groupe socialiste. Hé oui madame la sénatrice, j'ai son. Et j'ai parfois fait retirer de l'uniforme des policiers, des gendarmes parce qu'ils doivent être exemplaires. Mais je ne serai jamais dans la démagogie, comme vous l'êtes madame la sénatrice, qui consiste. À comparer de manière équitable. Les violences de la police, je mets des guillemets des violences des casseurs. Parce que quand on met un trait égal quand on dit violence policière et José casseurs, on a l'impression finalement, tout ça est un conflit. Et que il y a des 2 côtés des gens qui mériterait effectivement l'égalité le Parti socialiste a oublié Clémenceau le Parti socialiste a oublié monsieur Cazeneuve le Parti socialiste Monsieur Badinter. Je me rappelle pas du maintien de l'ordre évidemment que vous avez mis en place vous-même que nous on a corrigé parce que c'est nous qui avons présenté au Conseil d'État schéma le match à Lens qui a été validé, madame la sénatrice en disant dit oui mais. Vous répondez au vieil adage de ma grand-mère qui était femme de mineur ma grand-mère me disait quand on dit oui mais c'est que la phrase. Bien sûr, bien sûr, on a tous compris que vous aviez un grand problème ennuis avec la NUPES pour soutenir les forces de l'ordre et chacun le voit, chacun le voit dans l'opinion de la République. Les policiers ne veulent pas de lui mais oui il y a de l'exigence mais ils veulent du soutien parce que ce sont des femmes et des hommes. Fort mal payé, malheureusement qui protège nos concitoyens et comme hier, ils l'ont démontré, permet à chacun de manifester dans de bonnes ce conditions le procès que vous faites, madame la sénatrice. Et là encore, je suis prêt à répondre assez longuement quand il voudra au président de la commission des lois, aux policiers de la République n'est pas digne d'un grand parti de gouvernement comme le vôtre. Monsieur le Monsieur le président. Je voudrais dire au Ministre de l'Intérieur 4 Ministre de l'Intérieur, ce n'est pas seulement être le Ministre de la police. Mais vous êtes en charge de la paix civile, donc vous devez non seulement défendre les policiers et les gendarmes et vous devez veiller au respect de l'État de droit. C'est ce que les Français attendre le respect de l'ordre mais dans la justice et puisque vous vous référez à des grands Ministre de l'Intérieur de gauche, permettez-moi de me référer à Pierre Joxe avec qui j'ai eu l'honneur de travailler au ministère de l'Intérieur. D'une part plan quinquennal de modernisation de la police d'autre part, création de la direction de la formation. Instauration du code de déontologie leur maintenant. Déclaration des droits de l'homme dans les commissariats. Voilà le modèle que vous devriez suivre. La parole est à notre collègue Daniel crémier pour le groupe Les Républicains. Ce président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les négociations européennes sont totalement défavorable à l'énergie nucléaire, c'est grave. C'était Energie-n'a été intégré à la taxonomie verte qu'au prix de conditions drastiques pour preuve. Les autorisations délivrées après 2042, 1045 en sont exclus. De même que les activités de maintenance et du cycle. Aujourd'hui la directive ENR 3 et le règlement industrie à zéro émission l'exclut également la réforme du marché. L'électricité est toujours en attente. C'est un non-sens pour le climat, car cette énergie n'émet que 6 grammes de CO2 par kWh. Selon l'étude de l'Ademe. C'est un non-sens pour l'industrie car la moitié des États membres disposent d'un parc nucléaire et un quart envisagent de nouveaux réacteurs, c'est un manque cruel de crédibilité car il est illusoire de décarboner 75% de l'hydrogène dans l'industrie ou 5% dans les transports sans source nucléaire, le gouvernement n'a pas conduit la politique à la hauteur des enjeux. C'est une faute, il aurait fallu négocier plus presque ossements plus fortement. Pour parvenir à un compromis admissible. Je rappelle d'ailleurs que le Sénat a tiré le signal d'alarme depuis longtemps à travers sa résolution de décembre 2021 sur la taxonomie verte et celle de mars 2022 sur le paquet. 55 c'est aussi un point d'alerte de son rapport transpartisan de juillet dernier. Monsieur le ministe que compte faire le gouvernement pour obtenir enfin satisfaction auprès de ses partenaires européens, y a-t-il encore un couple franco-allemand, il faut garantir à l'énergie, l'hydrogène nucléaire une complète neutralité technologique. Il en va de notre souveraineté énergétique et nous faisons de nos engagements climatiques. Pour vous répondent la parole économiste délégué en charge de l'industrie. Monsieur Lescure. pour l'engagement que vous avez eu depuis maintenant de nombreuses années, vous avez fait référence à certaines dispositions adoptées par le Sénat et mais plus récemment aussi en tant que rapporteur du projet de loi présenté par le gouvernement pour l'accélérer la mise en oeuvre des projets nucléaires que nous avons qui a été voté par cette assemblée par plus de 9 sénateurs sur 10 ce même projet de loi a été votée la semaine dernière par l'Assemblée. Ça. Cinq donc 75% des députés l'ont voté, montrant que l'Union nationale derrière le nucléaire, ce qui n'a pas été tout le temps le cas est aujourd'hui de mise en France cette union nationale. Elle nous permet de porter haut la voix de la France en Europe et de négocier. Vous l'avez dit avec difficulté l'engagement de l'Europe qui doit reconnaître le nucléaire comme une des sources d'énergie de l'avenir, vous le savez, la France ne fait pas tout toute seule en Europe, nous sommes 27 aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous réponds et non pas la ministre de la transition énergétique, qui était à Bruxelles hier et qui est à Berlin. Aujourd'hui, nous continuons ces négociations hier la ministre était avec ce qu'on appelle l'Alliance du nucléaire. 11 pays qui en Europe, défendent le nucléaire comme une source d'avenir qui sont aujourd'hui allié avec la France et qui sont prêtes à bloquer un certain nombre de discussions pour s'assurer que nucléaire fera partie du futur. Nous avons, vous avez parlé du couple franco-allemand qui dirais un tango un peu difficile à mener avec eux c'est vrai ils ont la conviction que l'hydrogène de demain sera importé et renouvelable. Nous sommes convaincus que l'hydrogène de demain, il sera produit en France est nucléaire. Nous devons trouver un compromis. Nous avons besoin d'énormément d'hydrogène pour décarboner l'industrie. Nous allons continuer à travailler dans ce sens et merci, franchement, sincèrement au Sénat et à l'Assemblée nationale de son soutien du gouvernement dans ce combat, dont il faut le reconnaître qu'il est difficile mais que nous allons mener et gagner. Merci. Aujourd'hui, la France souffre, on est en pleine crise énergétique au niveau des familles, au niveau des collectivités, des entreprises. Aujourd'hui on est devant un défi. Le niveau de l'emploi, nous ne réussirons de nouveau nucléaire que si nous interventions des jeunes, nous sommes dans le doute. Monsieur le Ministre, il y a un véritable défi, celui de l'article 194 du fonctionnement de l'Union européenne qui précise que chaque État membre a le droit de choisir son mix énergétique. Aujourd'hui la France est bafoué. La France n'est plus respecté au niveau de ses choix stratégiques pour notre pays. La La parole est à notre collègue Jean agrée pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole. monsieur le président, Mesdames, et messieurs les Ministres, ma question s'adresse à Ministre à Madame, la ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur depuis le début de ce mouvement social hostile à la réforme des retraites. Des dizaines de lycées et d'universités ont été paralysés. Même la faculté d'Assas pourtant réputée la plus conservatrice de France a été également bloqué et cela pour la première fois de son histoire. Votre gouvernement aura incontestablement réussi quelque chose dans cette douloureuse réforme faire par un lire d'envie Dany le. la grève le blocage la manifestation deviendra deviendrait presque un rite initiatique dans notre pays. Chaque génération veut sa grande mobilisation chaque génération veut son Mai 68. Au-delà de ces manifestations, se cache la précarité, le mal-être des étudiants. C'est pourquoi Madame la Ministre mes interrogations sont multiples. Que comptez-vous faire pour empêcher une minorité de bloquer la majorité. Que comptez-vous faire pour que les examens se déroule dans de bonnes conditions, que comptez-vous faire pour les étudiants qui attendent des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien. Pour vous répondre. La parole est à la ministre de l'enseignement supérieur et de la région. Serge Madame Retailleau. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Jean agrée. Alors tout d'abord, effectivement, vous l'avez dit, une partie des universités sont bloquées aujourd'hui quelques dizaines sur les 200 universités et écoles avec quelques campus mais aussi des universités qui connaissent des blocages avant les manifestations et qui sont très relayée. Je voudrais signaler et dire, redire, mais vous le savez, que l'université est aussi d'abord un lieu d'émancipation et d'échanges mais aussi de confrontation des idées je voudrais et on le partage. Si les jeunes n'exprimait pas leurs idées, je pense qu'on craindrait pour notre démocratie. Pour autant, et pour autant le côté de blocage même temporaire d'empêcher les étudiants d'accéder à leurs études. Ce n'est pas le acceptable mais il faut le savoir, ce n'est pas l'apanage uniquement des étudiants. Je voudrais saluer la gestion du blocage à travers les recteurs et les préfets des régions et au travers de de la gestion par les présidents d'université. Alors cela m'amène à répondre à vos différentes questions et merci parce que aujourd'hui effectivement la précarité d'étudiants, les étudiants parle de beaucoup de choses dans les revendications et en particulier de leurs conditions d'études. Et je vous annonce donc aujourd'hui après des concertations que nous menons depuis le 7 octobre au niveau national et au niveau territorial avec l'ensemble des acteurs. Le gouvernement est sur la feuille de route du président de la République a débloqué un demi-milliard d'euros, 500 millions d'euros pour répondre à la vie étudiante à la gestion des bourses étudiants dès la rentrée 2023, mais aussi à la pérennisation du repas à un euro pour tous les boursiers et tous les étudiants précaires et d'autres mesures sur la vie étudiante, notre gouvernement, le président de la République et sur la feuille de route de madame, la Première ministre travaille pour donner des conditions des bonnes conditions à tous nos étudiants et ce que ce que nous allons faire dès la rentrée 2023. C'était un des dispositifs et des mesures historique avec une augmentation d'environ 20% sur les bourses de nos étudiants et sur les conditions de vie de nos étudiants, voilà la réponse que je peux vous faire aujourd'hui. Monsieur Oui très bien merci Madame la Ministre je pense. Que cette annonce régira les les bancs de ne de du Sénat, que ça soit des bandes de droite ou de la gauche puisque ce sont des demandes que nous faisons de depuis très longtemps l'augmentation des bourses dans une semaine nous proposerons avec mon collègue et ami Pierre-Antoine Levi. Une proposition de loi notamment sur les repas étudiants à tarifs modérés dans les zones rurales, les zones de montagne et aussi dans les petites villes, donc nous espérons que dans ces 500 millions, vous pourrez intégrer une partie du conventionnement avec les Crous en tout cas nous sommes vraiment très heureux de ces annonces qui, j'espère. Contribuera à atténuer la précarité et le mal-être étudiant même si ce n'est jamais assez. On peut se réjouir, au moins aujourd'hui de cette bonne nouvelle. Merci. La parole est à notre collègue Alain Cadec pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Et de la souveraineté alimentaire. Monsieur le Ministre, la France gronde. Et les marins-pêcheurs sont en colère. À une période où le prix du gasoil ne cesse d'augmenter. Après un plan de sortie de flotte qui pénalisent notre capacité de pêche. Après la proposition de la Commission européenne d'interdire les arts traînants c'est-à-dire chalut et drague dans les aires marines protégées, voilà que le Conseil d'État saisi par trois associations vous ordonne de fermer des zones de pêche dans le Golfe de Gascogne. Afin de protéger les dauphins dont la mortalité serait. Due à des captures accidentelles. Cela fait beaucoup. Je dirais même beaucoup trop. En effet si on additionne ces mesures, autant dire clairement qu'on abandonne l'idée de préserver une activité nécessaire à ce que tout le monde souhaite. Une relative souveraineté alimentaire. Le plan de sortie de flotte augmente encore un peu plus notre dépendance aux importations alors que nous en sommes déjà 70% de produits de la mer importés. Par ailleurs s'agissant de la fin programmée par les ONG et la Commission européenne des arts traînants la conséquence de cette mesure sera la disparition pure et simple de la pêche côtière. Plus de poisson, plus de poisson frais sur les étals plus de coquilles Saint-Jacques. Par exemple dans la gestion exemplaire. Il vous fait sourire la coquille. En tous les cas, sa gestion est exemplaire par la préservation de sa ressource. Ces décisions ubuesques vont nous condamner à importer davantage et à consommer de prendre des produits surgelés. C'est inacceptable, s'agissant des mesures de protection des cétacés, il existe déjà des dispositifs de dissuasion acoustique pour ces espèces dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Précisons au passage que les populations de dauphins sont en augmentation constante. Alors Monsieur le Ministre que comptez-vous faire face à ce déferlement de contraintes et d'interdiction qui à terme condamnera une activité porteuse d'emplois qui n'a jamais été aussi encadrer et aussi vertueuses. Pour vous répondre. La parole est à au ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Monsieur puisque comme vous le savez ou quoi mais il vous l'a peut-être dit Hervé Berville, elle est en déplacement. Lui même auprès des pêcheurs en Vendée. D'abord vous faire part, comme vous l'avez dit de la vous avez évoqué la colère des pêcheurs, elle est fort légitime devant une décision une proposition de la Commission européenne qui vise à interdire certaines techniques de pêche dans des aires maritimes protégées et qui s'apparente à un coup de massue, elle balaye cette décision ou cette proposition d'un revers de main tous les efforts qui ont pourtant montré leur capacité à être productif pour à la fois combiner les effets, les nécessités d'activité économique mais aussi la préservation des habitats marins. Le gouvernement a annoncé dès le 8 mars au Sénat c'était ici donc l'opposition de la France à ce texte et nous sommes les premiers à l'avoir fait, nous sommes désormais rejoints par un certain nombre de pays, l'important c'est d'avoir une coalition pour faire face et donner pièce à cette proposition 2ème élément c'est ce que nous faisons pour essayer donner aussi une perspective à la filière à la filière pêche et aux pêcheurs. Le président le la République et la Première ministre ont rappelé lors du salon de l'agriculture ils en place d'un fonds de 130 millions d'euros pour le secteur avec les aides carburants à la fin de l'année dernière, à Bruxelles, le gouvernement par la voix d'Hervé Berville a défendu face à la commission toutes les façades maritimes françaises pour maintenir les quotas de pêche et les rendent pluriannuelle pour donner enfin de la visibilité aux pêcheurs et nous soutiendrons la réduction de la dépendance au gasoil des navires de pêche et c'est ce que nous entendons faire enfin je le dis, c'est une filière qui est une filière clé, vous l'avez rappelé monsieur le sénateur, nous croyons comme vous dans cette filière qui fait partie aussi de l'identité française. La pêche maritime française est indispensable, indispensable aussi pour notre souveraineté. C'est donc sur ce chemin-là que nous essayons d'avancer à la fois face à des décisions de la commission qui paraissent incompréhensibles et à la fleur au rang des plans de soutien qui sont portés par le ministre Hervé Berville et qui est tout à fait aux côtés des pêcheurs malgré les difficultés que nous rencontrons, merci. La parole est maintenant notre collègue Thierry Cozic pour le groupe socialiste. Le le ministère. Merci monsieur le président, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et j'y associe. Mon collègue Rachid Temal. Depuis l'an dernier, l'inflation dans finit plus de de ne plus finir. Les prix des produits alimentaires ont grimpé de 14,5% en un an et une nouvelle hausse de 10% est à prévoir ces 2 prochains mois. Ce chiffre est en effet le plus élevé depuis 1985. Face à cela, quelle réponse vous apportez aux Français. Vous demandez aux enseignes de pratiquer pendant 3 mois je cite les prix les plus bas possibles sur un ensemble de produits leur choix. Je suis sceptique quant à la crédibilité accordée à ce genre de déclaration qui qui qui traduisent plus un voeu pieux que l'institution d'une mesure concrète. Cette volonté de rien imposer aux distributeurs est incompréhensible. Car, de l'aveu même de la BCE. Une grande partie de l'inflation serait tirée par la volonté des entreprises de sauvegarder leurs marges afin de maintenir leurs profits. Le candidat Macron nous parler de mettre en place pour les ménages les plus modestes. Un chèque alimentaire, ma question est donc simple. Quels engagements comptez-vous prendre devant la représentation nationale afin de donner un cap lisible et clair pour nos concitoyens, un cap qui ne soit pas l'otage de The revirements incessants et vos renoncements permanents, un cap que vous devez à nos concitoyens, tant la situation est difficile pour les plus précaires d'entre eux. Pour vous répondent, la parole est à la ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur. Czig vous parler de revirement quel revirement. Quel revirement quand depuis octobre 2021. Le président de la République Jean Castex à l'époque. Élisabeth Borne engage 110 milliards d'euros pour soutenir les factures d'électricité de nos concitoyens. Pas un pays européen n'a autant soutenu le pouvoir d'achat. Mais si on ne peut être en désaccord sur beaucoup de choses mais pas là-dessus 110 milliards d'euros, c'est pas de la flûte, monsieur, je vous réponds, il y a au moins le respect de m'écouter, ce serait sympathique. 110 milliards d'euros. Ça se vérifie 46 milliards 46 milliards juste sur l'année 2023 pour accompagner les factures d'énergie. Et alors excuse moi et j'ai encore la liberté de regarder ou je veux oui merci. Non. Suivez. Je vous remercie. Donc, ce gouvernement n'a jamais eu de revirement en matière de soutien au pouvoir d'achat, vous le savez très bien et le soutien il est massif et d'ailleurs vous l'avez voté ici. Aux côtés des Français. Ensuite vous critiquez avec. Force le trimestre anti-inflation que nous avons mis en place avec la grande distribution, c'est la première fois et vous le savez pour connaître ces sujets monsieur le sénateur. Que la grande distribution de façon unanime s'engage sur trois mois. Vous savez très bien qu'en général les promotions. Ces deux à 15 jours de promotion 3ème engagement au-delà d'être un engagement rapide et collective cet engagement il est juste. Ils prennent sur leurs marges pour assurer que les prix n'augmentent pas avec Bruno Lemaire, nous avons donc beaucoup travaillé avec eux durant 3 mois ce trimestre anti-inflation propose des centaines de produits à nos compatriotes. La direction générale de la répression des fraudes et de la concurrence surveille d'ailleurs aux côtés des distributeurs que les marges sont bien prises les les efforts sont bien faits sur les marges des distributeurs et nous avons appelé avec Bruno Lemaire à ce que il y ait possiblement une nouvelle négociation pour faire baisser les prix. S'il continue à baisser le prix des matières premières au printemps, au mois de mai avec les industriels alors aucun revirement de la volonté de la détermination et une inflation qui au global demeure l'une des plus faibles d'Europe. Je vous remercie Madame la Ministre, les Français ont besoin de stabilité, chèque alimentaire abandonner panier anti-inflation abandonné à la fin, je crains que ce soient les Français qui soit abandonnées avec vos dispositif. Monter comme une usine à gaz. C'est 50 nuances de prix. Dans un panier percé, avec l'abandon du panier inflation vous placer le pays dans les mains de la grande distribution dont les marges ne faiblissent pas. Tout en faisant passer ces dernières comme les principaux acteurs de la lutte contre la vie chère. La République en marche se mue en la République en marge. Bon faut qu'on pourrait en rire si à la fin, ce n'était pas le consommateur qui payait tous vos revirement. La parole est à notre collègue Corinne Imbert. Pour le groupe les républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé et de la prévention et j'associe à cette question mais 2 collègues Marie-Pierre Richer et Bruno Belin. Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interroger sur le projet de décret relatif aux conditions de transfert. Et de regroupement des officines de pharmacies qui prévoirait de définir des territoires fragiles, au sein desquels l'accès aux médicaments pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante, alors même que nous savons que 99,5% de la population française habite à moins de 15 minutes d'une pharmacie. Ce projet de décret proposerait de critères pour sélectionner ses territoires sachant que les pharmacies exploitées par un seul pharmacien titulaire de plus de 65 ans seraient exclus du calcul comme si aujourd'hui ils ne remplissaient pas leurs missions. Alors pourquoi les écarté sauf à vouloir peut être récupérer la licence pour faciliter un transfert une installation dans une zone plus peuplé. Monsieur le Ministre où en est ce projet de décret dit territoires fragiles en matière de transfert d'officine jusqu'à quel niveau. Le pouvoir des agences régionales de santé sera-t-il élargi en matière d'autorisation de transfert et de regroupements d'officines et surtout, Monsieur le Ministre, que faites-vous de l'aménagement du territoire et de la prise en compte du maillage existant. Pour vous répondre. La parole est au ministre de la Santé. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Hein ben. 21.021 1000 officines couvre actuellement le le territoire national. Ce sont souvent dans certains territoires le 1er recours à un professionnel de santé, ce sont les plus visibles et je tiens vraiment ici à les saluer ils tiennent cette première ligne dans de nombreux territoires et ils ont assuré leur fonction pendant la crise sanitaire et et encore de façon quotidienne. Pour autant, même si comme vous le dites, l'immense majorité du territoire est couvert pour autant il existe encore des territoires je pense à la Corse, je pense à la Guyane où 18% de nos concitoyens sont trop loin d'une pharmacie, c'est un peu le cas aussi sur certains territoires dans le Grand-Est, que je connais bien mais aussi dans le dans le Centre-Val de Loire. Donc la situation n'est pas totalement satisfaisante même si, globalement, on a une, une vision tout à fait correct. Alors c'est l'ordonnance du 3 janvier 2018 qui propose donc ce décret et qui propose de faire une adaptation, territoire par territoire. C'est tout l'esprit de la réforme du système de santé que nous portons aujourd'hui c'est aussi tout l'esprit des CNR santé qui ont été mis en place dans une logique de dialogue territorial avec les professionnels de santé concernés avec les élus et avec les citoyens. Dans cette logique. Nous sommes encore en train d'élaborer des critères pour que ce décret soit le plus opérationnel possible. Il y a des critères de distance mais il y a également des critères populationnelle en particulier des territoires où il y aurait beaucoup de personnes âgées qui n'aurait pas de moyen de se déplacer. C'est donc vraiment du travail de dentellière, territoire par territoire, qu'il va falloir faire, c'est pour ça que ce décret. Est bientôt fini. Il est encore en cours d'élaboration. On ne s'interdit rien et je discute avec les représentants des pharmaciens pour que vraiment il puisse répondre à ces citoyens qui sont encore trop loin d'une réponse de pharmacie. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre pour. Le dommage que vous avez rendu au aux pharmaciens d'officine qui effectivement font partie des professionnels de santé en première ligne. Vous avez cité 28.000 officines ça fait moins 4000 officines depuis quelques années, vous n'y êtes pour rien mais ça peut être un état, Le problème c'est que il y a une contradiction entre. Cette volonté ce qui motiverait la rédaction de ce décret pour répondre à quelques situations que vous avez exposés et ses conséquences qui conduiront à déstabiliser ce qui est aujourd'hui un exemple en matière d'aménagement du territoire les officines de pharmacie représente une vraie colonne vertébrale en matière d'accès aux soins en matière d'aménagement d'aménagement du territoire et vous savez et vous ne l'ignorez pas, et c'est ce décret qui ne devrait pas fragiliser l'existant. Aujourd'hui de nombreux Français vivent dans des déserts médicaux. Je vous en supplie Monsieur Ministre il devient urgent de ne pas y ajouter des déserts pharmaceutiques si vous déstabiliser de réseau, vous allez. Vous allez comment dire nuire au au patients et favoriser non seulement peut-être des gros investisseurs. Mais s'il vous plaît, monsieur le président. Une fois de plus vous avez sacrifié l'aménagement du territoire et du et évidemment le monde rural et ça ça ne serait pas acceptable, je vous remercie. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le législateur a confié à La Poste, 4 missions de service public dont la contribution à l'aménagement du territoire. Celle-ci se traduit par l'obligation de maintenir un réseau de 17.000 points de contact, ce qui garantit une densité du réseau postal spécifiquement française. Le 15 février dernier, l'État l'AMF et la Poste ont signé le 6ème contrat de présence postale territoriale pour la période 2023 2025. Celui-ci fixe le cadre permettant à la Poste de contribuer à la mission d'aménagement du territoire. Il prévoit les règles d'adaptation de son réseau et de gestion du fonds de péréquation territoriale. D'un montant annuel de 174 millions d'euros, il doit bénéficier prioritairement aux zones qui en ont le plus besoin. Face à une fréquentation en chute libre des bureaux de poste. La mutualisation des réseaux territoriaux de la Poste et de l'État est une condition de survie selon le contrat. Mais en 2021. Le coût du maintien d'un maillage territorial fin du service postal a été évalué par l'Arcep, à 348 millions d'euros tandis que la compensation reçue n'a été que de la moitié. Cette sous-compensation risque d'être très pénalisante en ne permettront plus d'accomplir les investissements utiles. Je tiens à préciser que la gestion de ses crédits et largement décentralisés et déconcentrés pour un pilotage réactif et Agile des projets conçus au plus près du terrain, par l'intermédiaire des CD PPT. Alors Monsieur le Ministre, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour remédier à cette sous-compensation et faire que la qualité, l'offre de service, ainsi que l'accessibilité postal soit une réalité dans nos territoires. Je vous remercie. Pour vous répondre. La parole est au ministre délégué en charge.

L'état l'AMF et la Poste ont signé le 6ème contrat de présente possède qui tire les enseignements du contrat précédent ainsi que du rapport que vous avez commis avec vos collègues, Pierre Louÿs et Rémi Cardon avec Bruno Lemaire Gabriel Attal et Dominique Faure nous avons veillé à ce que ce contrat fasse figurer 5 priorités, d'abord le maintien de la présence territoriale de la Poste dans un contexte, vous l'avez dit de baisse très marquée du, du trafic dans les bureaux de poste en accompagnement du déploiement du réseau France service sur lequel veille attentivement Stanislas Guerini sont donc 17.000 points de contact qui seront maintenus sur le territoire d'une dotation de 174 millions d'euros, une plus grande accessibilité horaires des bureaux de poste notamment le week-end et lors des événements locaux, le renforcement des actions de médiation sociale et numérique à destination des populations vulnérables, j'y suis particulièrement attentif et puis l'amélioration de la gouvernance des commissions départementales pour une meilleure utilisation du fonds de péréquation. Il faut rappeler que toutes ces actions financées sur ce contrat. Vont bénéficier prioritairement aux territoires ruraux au territoire de la politique de la ville aux zones de montagne et aux territoires ultramarins et puis rappelez pour répondre à votre question que le gouvernement s'est engagé à ce que ce soutien se poursuivent par une dotation qui sera discuté dans le cas du projet de loi de finances 2024 2025 et dont vous aurez à débattre, vous le voyez, Monsieur le Sénateur, sous l'autorité de la Première ministre, le gouvernement extrêmement vigilants à ce que la Poste puisse remplir dans les meilleures conditions, sa mission de service public. Merci monsieur le président. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse qui me laisse beaucoup d'espoir. Vous comprendrez bien que la sous-compensation et l'augmentation des dépenses obligatoires aujourd'hui assèche le système. Sans ne rien modifier de façon favorable on rend incohérent. Les discours et les actes. Alors pour redevenir cohérent. Je vous donne l'occasion, Monsieur le Ministre, d'améliorer la sous-compensation pour faire en sorte que les Français aient confiance en vous. Merci. Informé, le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion. Du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. Merci madame, la Première ministre. Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues, nos prochaines questions d'actualité auront lieu le 5 avril à 15h. Je vais lever la séance est notre prochaine séance aura lieu le mardi 4 avril, 2023 9h 30 pour les questions orales. La séance est levée.